La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Je rappelle que la discussion générale a été close. Nous passons à la discussion du texte

Lors de l'examen de la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire du 11 mai dernier, le Sénat avait adopté l'amendement de notre collègue Véronique Guillotin, visant à renforcer les garanties contre tout effet d'aubaine concernant les produits sanitaires de première nécessité au moment d'une crise sanitaire. Il s'agissait de permettre une meilleure publicité des prix contrôlés, auprès des consommateurs, mais également des professionnels.

Mis en place le 23 mars dernier, l'état d'urgence sanitaire avait méthodiquement organisé le placement en quarantaine de nos libertés individuelles, fondamentales et politiques. Face à la crise liée au Covid-19, nous avions accepté cet état de fait, tout en dénonçant les possibles dérives d'un tel droit d'exception. Force est de constater, hélas, que nos craintes étaient fondées : alors que le Gouvernement s'apprête à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet prochain, il estime également nécessaire de s'approprier certains de ses outils jusqu'au 30 octobre ! Si cet article était adopté, en cas d'un risque nouveau de propagation du virus, le Premier ministre et le préfet se verraient notamment attribuer le droit de réguler la circulation des individus, d'aménager le fonctionnement des établissements recevant du public et, surtout, de réglementer la tenue des rassemblements. Une telle volonté est incompréhensible ! Si l'exécutif demande la fin de l'état d'urgence, c'est qu'il estime que la crise sanitaire est sous contrôle. pour quelles raisons souhaite-t-il entraver la capacité de nos concitoyens à se réunir et à manifester ? Entre droit d'exception et droit commun, le Gouvernement veut désormais définir une troisième voie transitoire, dans laquelle le premier se fondrait dans le second. Une telle situation n'est pas souhaitable. Avec la fin de l'urgence sanitaire, devrait arriver le déconfinement de nos droits et libertés. L'exécutif ne saurait se livrer à une gouvernance solitaire par décrets, venant restreindre et réguler nos moindres faits et gestes. Très bien

de notre président de la commission des lois- elle est grande -, toute la détermination des membres de cette même commission des lois- elle n'est pas moins grande -pour trouver un chemin qui, pour ne pas être nouveau, était très étroit, nous permettant de ne pas rejeter le texte.

une singularité française qu'il conviendra d'étudier- pas ce soir, mais à l'avenir. Nous avons eu le confinement le plus rugueux, le plus dur, le plus long. Nous avons sans doute eu, de toutes les économies occidentales et européennes, l'arrêt le plus brutal. Enfin, nous avons eu un état de droit parmi les plus contraints : le Parlement a travaillé difficilement, la justice s'est presque interrompue, et il y a eu un transfert massif des pouvoirs vers l'exécutif.

Je ne pensais pas avoir si bien dit, monsieur le ministre ! Le « en même temps et tout à la fois » que vous nous proposez ne convient pas, d'où cette demande, par le groupe socialiste et républicain,

dans sa substance, tout en consentant à sortir formellement du cadre de la loi du 23 mars 2020, et ce pour une durée de quatre mois minimum, qui pourrait donc être

il faut le dire ». Or les modifications que vous avez proposées et fait voter par la majorité de la commission des lois ne permettent pas, selon nous, de sortir de l'ambiguïté que vous dénoncez. Elles sont elles-mêmes,

de réglementation pourra parfaitement masquer une forme d'interdiction. Comme vous l'indiquiez, ou nous sommes dans un état d'urgence, ou nous ne le sommes pas. L'attitude claire, courageuse, pour faire respecter les libertés publiques et les pouvoirs du Parlement est donc celle du rejet de ce texte, tout particulièrement de son article 1. Comment ne pas remarquer que la prolongation de mesures d'exception- le texte le texte de la commission s'inscrit, malgré tout, dans ce cadre jusqu'au 30 octobre -diminue encore, par rapport à l'état d'urgence sanitaire, classique ou d'exception, le pouvoir d'intervention

En effet, cet article prolonge des mesures restrictives des libertés fondamentales et des droits qui ont été mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; il vient ainsi brouiller la frontière entre l'exception et le droit commun, avec tous les risques que cela comporte pour l'État de droit. Alors que la population est appelée à voter pour le second tour des municipales, que les activités économiques reprennent- et c'est tant mieux -et que la situation sanitaire continue de s'améliorer- et c'est aussi tant mieux -, la proposition du Gouvernement de créer ce nouveau régime dérogatoire est à la fois disproportionnée et inutile. En effet, le droit existant, cela a déjà été expliqué à plusieurs reprises lors de nos débats, est largement suffisant pour gérer la situation sanitaire. Et, en cas de résurgence de l'épidémie, le Gouvernement et le Parlement auraient la capacité de prendre les mesures nécessaires, et cela en urgence. Certes, cela a été souligné, la commission des lois a limité fortement la portée de cet article en proposant de donner au Premier ministre le pouvoir de réglementer, plutôt que d'interdire. Cela atténue indéniablement les restrictions de libertés proposées par le texte.

de ce fait un entre-deux pour nous inutile. De plus, le contexte actuel doit nous amener à être plus que vigilants sur la question des restrictions apportées aux libertés ; je pense en particulier au droit de manifestation. Rappelons que le Conseil d'État a considéré la limitation de ce droit fondamental prise dans le cadre de l'état d'urgence comme une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté de manifester, alors que, après plusieurs mois de limitation des libertés publiques et à l'heure où s'organisent les débats sur le monde d'après, les citoyens ressentent légitimement le besoin d'exprimer collectivement leurs idées, et cela en toute liberté. Quel

je considère qu'un texte de sortie de l'état d'urgence sanitaire qui reproduit les mesures les plus importantes de l'état d'urgence sanitaire est un texte de prorogation de l'état d'urgence sanitaire ! En outre, je veux bien admettre que, comme l'indiquait

plus. Je ne vous demanderai pas de retirer vos amendements ; ils sont pour vous le moyen de marquer très clairement une position politique. ma part, j'essaie d'être pragmatique et d'apporter des réponses. C'est notre rôle à nous, sénateurs, non pas d'adopter une position qui soit exclusivement politique, mais de chercher des solutions qui n'exposent pas les libertés

ce qu'elle est et vous entendez les appels au secours de nos collègues de Guyane et des territoires ultramarins, qui disent le manque de masques, d'équipements, le besoin de médecins,

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Nous accueillions avec soulagement, mais prudence, cette nouvelle, qui laissait présager un prochain retour à la normale. Dans ces conditions, il semble légitime que l'état d'urgence sanitaire, instituée par la loi du 23 mars 2020, prenne fin. Nous tenons donc à pointer du doigt l'incohérence du Gouvernement, qui souhaite ici créer un droit hybride entre le droit commun et le droit d'exception en vigueur pendant l'épidémie. Monsieur le ministre, si vous estimez que la pandémie est suffisamment sous contrôle pour que nous puissions nous passer de l'état d'urgence sanitaire, agissez en conséquence Que des réglementations soient conservées un temps, notamment en matière de port du masque ou de respect des gestes barrières dans les transports en commun, nous l'entendons parfaitement. Ces précautions nous semblent tout à fait raisonnables. Mais il nous paraît excessif de conférer ces prérogatives au Premier ministre. Une telle mesure, attentatoire à l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la liberté de circulation, est disproportionnée à l'heure où l'exécutif souhaite assurer une transition vers la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, par le présent amendement, nous demandons la suppression de l'alinéa 2 de l'article 1. Le virus est toujours présent, mais il est latent. Nous sommes donc favorables à ce que des précautions soient de mise, mais sans disproportion. L'amendement Cet amendement du Gouvernement vise à préciser la portée des notions retenues au premier alinéa de l'article 1, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois. La faculté générale de réglementer la circulation des personnes et des véhicules doit permettre d'intégrer, le cas échéant, des mesures de restriction de la circulation des personnes ou des véhicules au-delà d'un certain périmètre d'un certain périmètre géographique, sans donner pour autant la possibilité de prendre des mesures assimilables à des interdictions de sortie du domicile, comme le prévoyait l'état d'urgence C'est ce qui permettrait d'ailleurs, en cas de cluster ou, plus largement, en cas de résurgence de l'épidémie, de limiter la circulation au-delà d'une zone, par exemple une ville,

que vous puissiez imposer le port du masque dans le métro, bien sûr, mais nous ne voulons pas que vous puissiez interdire un certain nombre de déplacements. Si vous devez le faire,

mesure ? Dès lors, pourquoi vouloir interdire ou retirer au Gouvernement la possibilité de limiter temporairement la circulation en dehors d'une zone d'activité du virus ? Quel usage considérez-vous que nous pourrions faire

Je reste cohérent

-et sans mettre en péril l'économie, à un degré tel que nous nous attendons tous à une vague de chômage dont les conséquences sociales et sanitaires, liées à la précarité, sont l'horizon des Français pour les années à venir. Bien sûr ! Si vous, ministre de la santé,

Ce pouvoir lui serait confié après la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet, et jusqu'au 30 octobre prochain en cas de rebond du nombre de contaminations liées au coronavirus. Ces dispositions pourraient notamment être appliquées aux monuments historiques, aux lieux de culte et aux restaurants. Une telle mesure semble disproportionnée et peu raisonnable au regard de la conjoncture économique. Les secteurs du tourisme et de la restauration ont été durement frappés par la crise liée au Covid-19. Leurs pertes s'élèvent aujourd'hui à plusieurs milliards d'euros. Il est vital que ces pans de l'économie puissent reprendre une activité normale dans les plus brefs délais.

La commission propose d'écrire que, « sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure », le Premier ministre peut « réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public Nous comprenons ainsi que le Premier ministre pourra réglementer tous les rassemblements mentionnés au quatrième alinéa, y compris, le cas échéant, pour les soumettre, non à autorisation préalable, comme c'est aujourd'hui le cas en vertu de l'état d'urgence sanitaire, mais à une simple déclaration préalable. Le préfet aurait dès lors la possibilité de les interdire en cas de troubles graves à l'ordre public, au sens de l'article L. 211-4, lequel inclut les risques sanitaires, comme l'a jugé le Conseil d'État dans son ordonnance du 13 juin dernier.

dans une zone de circulation de l'infection et qui souhaitent se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance de l'Hexagone ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage ne concluant pas à une recontamination par le Covid-19. Bien sûr, toutes les mesures doivent être prises pour protéger les citoyens qui, en raison de leur situation aux confins du territoire national, sont particulièrement vulnérables face à un risque épidémiologique.

À la veille des grandes vacances, nous nous interrogeons également sur la capacité actuelle de dépistage. Nous craignons que, faute de tests, beaucoup ne renoncent à leurs déplacements. Une telle entrave à la liberté d'aller et venir serait susceptible de porter atteinte au secteur touristique insulaire et d'infliger un grave manque à gagner aux compagnies aériennes. C'est pourquoi nous proposons

de se déplacer en avion, à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou d'une collectivité d'outre-mer. Mais cette rédaction est beaucoup trop large

cet alinéa est particulièrement révélateur du rôle que l'exécutif souhaite confier au Parlement dans le cadre de la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire. Alors que le Premier ministre serait habilité à légiférer par décret, le Parlement, lui, serait cantonné dans un rôle d'observateur, que l'on informe par courtoisie institutionnelle. Faut-il le rappeler ? C'est bien le Gouvernement qui est responsable politiquement devant le Sénat et l'Assemblée nationale, et c'est bien le Parlement qui a pour mission constitutionnelle de légiférer. Il n'est pas acceptable que les chambres soient réduites à un rôle d'enregistrement et d'habilitation de l'exécutif à légiférer par ordonnances ou par décrets.

il est urgent que les élus de la Nation et des territoires retrouvent leur capacité d'édicter les lois ! Quel

répressives, visant à garantir la sécurité de nos concitoyens pendant la crise sanitaire en sanctionnant le non-respect des règles édictées en vue de contrer la pandémie : le confinement, puis le port du masque et l'application des gestes barrières dans les transports en commun et les lieux publics.

si une augmentation du nombre de cas de Covid-19 est à déplorer. Les auteurs du présent amendement dénoncent la banalisation à laquelle s'adonne l'exécutif s'agissant de mesures coercitives et répressives et répressives : introduites dans notre législation en raison de la crise sanitaire, elles ne sauraient être utilisées en dehors du cadre dans lequel elles ont été édictées. Figurant à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, ces dispositions pénales n'ont pas vocation à voir leur champ d'application élargi.

par l'ensemble de nos concitoyens, mais peut-être encore plus par ceux de l'outre-mer. Dans les territoires insulaires, en effet, la suspension des moyens de transport a des conséquences beaucoup plus importantes qu'en métropole sur toutes les chaînes d'approvisionnement, et réguler la saturation des hôpitaux y est

de nouveau un amendement gouvernemental ... Quelque chose me dit que celui-ci peut passer

trois territoires, l'enjeu est donc de permettre la reprise normale des liaisons aériennes, ainsi que le retour progressif des touristes et des Ultramarins de l'Hexagone qui rentrent passer les grandes vacances dans leur famille, tout en maintenant des mesures de contrôle sanitaire pour empêcher l'importation du virus.

il est nécessaire de maintenir un contrôle sanitaire pendant les prochains mois, sous la forme de tests virologiques obligatoires pour les personnes souhaitant se rendre en outre-mer, afin de permettre la reprise du tourisme tout en protégeant la population. Il s'agit d'une demande très forte des territoires

au prétexte de l'épidémie de Covid-19. Vous avez ainsi autorisé les employeurs à imposer unilatéralement des jours de congé aux salariés et aux fonctionnaires, et les entreprises considérées comme « relevant de secteurs particulièrement nécessaires

Depuis trois mois, donc, les entreprises peuvent pleinement profiter du dérèglement du travail pour exploiter toujours plus les travailleuses et les travailleurs, Pourquoi le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ne prévoit-il pas aussi un retour à la normale pour les droits des salariés ? Pourquoi faudra-t-il attendre la fin décembre pour que soient rétablis le repos dominical et la liberté des jours de repos ? Hier, vous nous expliquiez que les dispositifs mis en place par le Gouvernement étaient justifiés par l'urgence de la pandémie et l'impossibilité pour les entreprises de travailler normalement. Aujourd'hui, à vous entendre, c'est la reprise économique qui justifierait de remettre en cause les règles essentielles de santé et de sécurité au travail. Demain, les risques d'une seconde ou d'une troisième vague de Covid-19 justifieront le maintien de ces dispositifs dérogatoires temporaires. Ainsi le Gouvernement transformera-t-il des dispositifs exceptionnels

ni entraîner, par un confinement généralisé, des conséquences dévastatrices sur le plan économique et social. Telle est la réflexion que nous devons mener, les uns et les autres, pour la faire converger.

Eh bien, pour une raison très simple. Si nous avions adopté votre article 1, reprenant textuellement trois dispositions essentielles de l'état d'urgence sanitaire, vous auriez disposé de moyens

de ne pas baisser la garde, en permettant au Gouvernement, dans cette période de sortie de l'état d'urgence sanitaire et non dans un an, de recourir à un instrument juridique qui s'est révélé,

donne au ministre de la santé, en réalité, les pleins pouvoirs. Je pense que le législateur n'a pas entendu lui donner de tels pouvoirs, mais, comme vous avez dû décider le confinement toutes affaires cessantes, avant même le vote de la loi

Au reste, Mme la ministre de l'outre-mer arrive demain en Guyane pour jouer les sapeurs-pompiers ... On ne peut que s'en réjouir, mais j'espère qu'elle apportera des réponses aux questions que nous avons posées voilà trois mois.

à la production de masques et de tests le Gouvernement a préféré le confinement, puis la mise en place d'un système informatique retraçant les chaînes de contamination au sein de la population.

Autant vous dire que l'article 2 de ce projet de loi n'est pas de nature à nous rassurer ... De fait, l'exécutif nous propose désormais d'allonger la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d'information mis en oeuvre pour lutter contre la pandémie. Or la conservation des données pose un sérieux problème de confidentialité et porte manifestement atteinte à la vie privée des Français. Pour seule assurance, le Gouvernement nous avait affirmé que la collecte et la conservation des données seraient strictement limitées à la durée de l'état d'urgence sanitaire. sanitaire. Si l'exécutif estime nécessaire que nous sortions le 10 juillet prochain de ce régime d'exception, pourquoi s'entête-t-il à vouloir conserver plus longtemps les informations liées à la pandémie ? J'ai bien peur que, une fois de plus, le Gouvernement ne fasse fausse route : pour réussir la sortie de l'urgence sanitaire et prévenir le risque d'une recrudescence du virus, il faudrait plutôt dépister que pister !

qui a été tranché, avec le soutien de plusieurs commissions de notre assemblée, dans le sens souhaité par le Gouvernement. Considérant que la priorité était donnée à la casse

à propos des données collectées par les brigades médicales. Les députés ont modifié cet article pour respecter cet accord. L'exploitation de leurs données personnelles à des fins épidémiologiques inquiète grandement nos concitoyens, qui craignent qu'elle ne soit dévoyée. Récemment, un chercheur a accusé l'application StopCovid de collecter des données plus importantes que ce qui était annoncé, notamment le nom des utilisateurs se situant à plus d'un mètre. Nous comprenons l'intérêt de la collecte de certaines données anonymisées pour la communauté scientifique. Cependant, l'examen du présent projet de loi se déroule dans des conditions de grande rapidité, qui ne nous paraissent pas satisfaisantes pour décider d'une nouvelle modification de ces règles quelques semaines

les données qui seront utilisées ne permettront pas d'identifier les personnes qui auront été atteintes de la maladie et serviront exclusivement à des enquêtes épidémiologiques.

d'enquêtes épidémiologiques. En revanche, pour ce qui concerne l'exploitation des données à des fins de dépistage, nous avons approuvé les restrictions apportées par l'Assemblée nationale au texte du Gouvernement. D'ailleurs, nous les aurions apportées nous-mêmes

Oui aux enquêtes épidémiologiques dépourvues de données permettant l'identification directe des personnes. Non à toute conservation de données personnelles à d'autres fins. J'émets donc un avis

et par l'autorité territoriale de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, donc par le Congrès- c'est le sens de l'amendement n° 6 -, soit,, après consultation des autorités locales-

que celles prévues » par le code de la santé publique. Cela pose un problème particulier, dès lors que ces collectivités ont été moins atteintes par le virus que le reste de la France. Pourquoi faudrait-il leur permettre de prendre des mesures plus contraignantes ?

L'amendement adopté en commission vise à supprimer la possibilité donnée au haut-commissaire de déroger aux mesures de quarantaine et d'isolement. On prive ainsi l'article 3, tel qu'il a été introduit à l'Assemblée nationale,

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ayant une compétence exclusive en matière de santé publique, revendiquent la possibilité de prendre, sur leur territoire, des mesures de quarantaine qui peuvent être différentes de celles qui sont prévues sur le territoire national. De même, leur stratégie de prévention doit pouvoir être différente. À

Les Polynésiens comme les Néo-Calédoniens estiment que les résultats qui ont été obtenus sur leur territoire sont précisément liés à la qualité du travail qu'ils estiment

il y a le texte et le contexte ... Nous nous sommes montrés responsables en votant, au mois de mars dernier, en faveur de la loi instaurant l'état d'urgence sanitaire. Nous ne pouvons néanmoins accepter que, une fois de plus, la gravité de la situation serve de prétexte pour faire entrer peu à peu un état d'exception dans le droit commun. Ce n'est pas la première fois que l'on nous ferait le coup, si vous me permettez l'expression. Ainsi, en 2017, vous avez opté pour l'intégration de mesures d'exception dans le droit commun, au travers de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

une tolérance inquiétante pour la tutelle de l'État, que l'on nous impose par petites touches. Mes chers collègues, il ne faut pas s'habituer à cette grammaire, qui ne surprend plus grand monde, y compris parmi nos concitoyens ... Bien évidemment, monsieur le ministre, il ne s'agit pas de minimiser la crise que nous traversons. Il s'agit de poser les bonnes questions. L'urgence commande-t-elle de prendre des mesures dont les conséquences à long terme ne peuvent pas toujours être mesurées ? Plutôt que de mal faire, n'est-il pas possible d'utiliser ce qui existe déjà, comme le code de la santé publique ? Mes chers collègues, je vous incite à méditer sur cette belle phrase d'André Breton : « On ne prend pas sans danger des libertés avec la liberté.